La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.

Mardi 11 janvier, le Conseil constitutionnel a évoqué en ces termes « la possibilité que [ ...] le Gouvernement élabore de nouvelles mesures d'organisation qui apparaîtraient rendues nécessaires par la crise sanitaire, afin de garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle ».

l'interdiction du recours au vote électronique et par correspondance, troisièmement, le rappel du droit de chacun de voter à l'urne en personne ou de faire une procuration. Pour rappel, le vote par correspondance est interdit en France depuis 1975, car il présente de trop nombreux risques de fraude. Le vote grâce à des machines électroniques est permis dans certaines communes depuis 1969, mais il n'a pas ramené les électeurs aux urnes, il a même suscité de la méfiance. La séquence politique majeure qui s'ouvre devant nous ne doit pas devenir un simulacre de démocratie. Madame la ministre, ne faites pas monter la peur dans ce pays pour balancer par la fenêtre nos bulletins de vote. Il ne s'agirait pas de décourager les électeurs, qui sont de moins en moins nombreux à chaque élection, au point que certains se sont crus autorisés d'en fabriquer dans les Ehpad marseillais ! Le suffrage vaccinal deviendrait le nouveau suffrage censitaire de ce régime, non universel, restreint et contrôlé : trois adjectifs qui conviennent à merveille à la politique gouvernementale actuelle. Pour balayer cet amendement, vous me rétorquerez qu'il est déjà satisfait par la Constitution ; je ne le crois pas. Pour rappel, le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a donné son accord pour l'instauration du passe sanitaire sous trois conditions

Mes chers collègues, si j'avais pensé qu'il y avait le moindre risque, j'aurais été le premier à proposer à la commission des lois un amendement de ce type. pas trop tard ! Pourquoi est-ce inutile ? Tout simplement parce que, de la même façon que pour le passe sanitaire, le passe vaccinal ne peut être exigé que dans des lieux limitativement énumérés par la loi elle-même.

dans les lieux qui sont prévus par la loi. Les bureaux de vote en sont absolument et radicalement exclus. Vous pouvez le répéter dans le texte sur tous les tons, vous n'ajouterez rien à la loi vous vous serez seulement fait plaisir. J'aimerais moi aussi vous faire plaisir, mais peut-être aurez-vous suffisamment de plaisir en sachant que votre intention est entièrement pourvue par le texte.

d'exercice de la démocratie. Pour ma part, je l'ignore totalement ! La démocratie est à la fois partout et nulle part. On exerce la démocratie et la citoyenneté partout où l'on se trouve

on nous avait promis que jamais on ne demanderait le passe sanitaire pour accéder à des meetings politiques ou des réunions publiques organisées à l'occasion de la campagne présidentielle.

qu'hypothétiques. En effet, à l'heure où la quatrième dose de vaccin est déjà évoquée, comment ne pas douter d'une stabilisation de la définition du schéma vaccinal complet, donc d'un recul incessant dans le temps du taux d'atteinte de couverture vaccinale à 80 % ? En outre, retenir comme critère l'accueil de moins de 10 000 patients dans les hôpitaux revient à conforter le Gouvernement, qui légifère pour pallier les carences de nos hôpitaux publics dont il est lui-même en grande partie à l'origine. Aussi, tous ces efforts, qui sont à saluer, qui accompagnent pour ainsi dire les cheminements du Gouvernement, ne remettent absolument pas en cause la logique sécuritaire et autoritaire en cours, laquelle devrait selon nous être renversée au profit d'une logique de gestion purement sanitaire et sociale de la crise.

de la commission des lois et de son rapporteur sur l'importante question des contrôles d'identité, lesquels restent, heureusement, une prérogative des forces de l'ordre. Espérons, mes chers collègues, que cela passe la rampe de la commission mixte paritaire.

Après la révolte et la résignation, c'est la lassitude qui pèsera sur la vie sociale de notre société pendant des mois et des années. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à ce projet de loi et nous nous opposons à l'article 1, malgré les modifications apportées

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je reste profondément guadeloupéenne et je représente ici les élus de la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve la population guadeloupéenne, compte tenu du taux de vaccination insuffisamment pris en compte par la population, même si l'on note une augmentation tant chez les personnels soignants que dans la population,

obliger toute la population à se vacciner et enchaîner les doses de rappel sous la menace d'une restriction des libertés permettrait de stopper l'épidémie et de diminuer la pression sur le système hospitalier, déjà bien malade. de la santé (OMS), qui affirme que des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin. Une fois de plus, l'exécutif semble céder à la panique. Marginaliser toute une partie de la population par l'instauration d'un passe vaccinal n'est pas une solution viable. Le ciblage et la protection des publics à risque devraient être privilégiés ; la pédagogie auprès des plus réfractaires devrait continuer ; l'utilisation des masques FFP2 devrait être renforcée et le traitement médical, développé. Le Gouvernement oublie de prendre en compte le caractère international de la lutte contre l'épidémie. Le variant delta venait d'Inde ; omicron vient d'Afrique du Sud. Dans ces pays, le taux de vaccination reste faible. Une levée des brevets est indispensable pour limiter la circulation des variants. Bien sûr, la France ne peut l'obtenir à elle seule, vu que nous ne fabriquons pas de vaccin

On combat, comme il est normal, les faux passes. Nous devrions aussi combattre la mauvaise utilisation du passe sanitaire, et demain vaccinal, dans notre pays. Les sanctions pénales prévues dans la loi sont très lourdes.

avec une profonde gratitude pour le travail remarquable et raisonnable qui a été accompli par nos commissions des lois et des affaires sociales. Aucun d'entre nous n'a voulu, n'a choisi, n'a provoqué une telle situation. Mais il nous appartient, tout en respectant les convictions des uns et des autres, et tout en saluant la qualité du débat dans cet hémicycle, de reconnaître que, face à cette difficulté, il convient d'accepter et d'adopter des mesures sans doute

Notre groupe considère que le passe vaccinal se rapproche de sa position, même si, d'une certaine façon, c'est une obligation vaccinale déguisée. Nous serons logiques,

encadrer et améliorer ce texte. J'aimerais remercier aussi notre président de groupe, Bruno Retailleau, qui a permis qu'une autre voix s'élève au sein des Républicains.

J'accuse le Gouvernement d'être responsable de la tension que vivent aujourd'hui nos concitoyens. Nous leur faisons vivre quelque chose d'insupportable : les jours de repos

La censure, le manque de transparence, les interdictions, les manipulations m'orientent vraiment vers le respect d'un principe de précaution. Je ne suis pas antivax. Pas du tout du tout ! Simplement, je suis, comme beaucoup d'autres citoyens, inquiète, et je réfléchis. Quand on est dans la juste décision, on est dans la transparence.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.

Oui, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la liberté est rognée par le passe vaccinal. Et celui-ci va impliquer la vaccination d'enfants, parce que 5 millions d'adultes n'ont pas été vaccinés et que notre hôpital est en

Quand on pratique l'art du mensonge, de la dissimulation et des contradictions, il ne faut pas s'étonner que la crédibilité de la parole publique soit atteinte.

Ce passe vaccinal est une obligation vaccinale déguisée, comme l'a dit Jean-Pierre Sueur. Les soignants sont obligés de se vacciner et, en cas

Monsieur le président, madame la ministre, la grande majorité de mon groupe votera l'article 1, qui institue le passe vaccinal. dire le sens de notre vote. Nous avons une arme, le vaccin. Ce n'est pas la seule arme, elle n'est pas parfaite, elle n'empêche pas les contaminations. Mais elle a un immense avantage, que j'ai rappelé plusieurs fois hier soir : elle prémunit contre les formes graves.

le nombre de lits de réanimation. La Cour des comptes a écrit que ces services ont été l'angle mort du Ségur de la santé. Enfin, nous sommes encore le pays où le taux de vaccination des plus fragiles est le plus faible.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

ne pouvons pas prendre de mesures générales consistant à prévoir qu'un vaccin devrait nécessairement être validé. Je comprends que nos compatriotes de l'étranger prennent les vaccins vaccins disponibles dans le pays où ils se trouvent ; j'espère d'ailleurs que ceux-ci produisent des effets bénéfiques. Mais je ne pense pas que le Parlement puisse être juge

Les règles posées en France ne seront pas forcément les mêmes que celles qui sont vigueur dans d'autres États de l'Union européenne. C'est purement factuel.

n'est pas du tout laxiste. Nous prévoyons qu'un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé détermine les exigences de vaccination qui seront requises en fonction des vaccins

Madame la ministre, nous

Alors que la France préside l'Union européenne, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dont le siège est à Strasbourg. En l'état, la France pourrait être maintes fois condamnée et contrainte de changer sa loi.

Selon cette jurisprudence, pour qu'une obligation vaccinale soit conforme à l'intérêt de sa population, il faut respecter quatre critères : que les maladies soient extrêmement graves et mortelles que les vaccins soient efficaces et les effets secondaires connus ; que les sanctions de la non-vaccination soient mesurées ; que le statut d'objecteur de conscience soit prévu. Si la Cour européenne des droits de l'homme devait se pencher demain sur la vaccination obligatoire contre la covid-19

Compte tenu des incertitudes et des risques pour l'avenir, il est de notre devoir d'admettre que la conscience de nos concitoyens peut être heurtée et de la protéger en créant

Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. » Comment avons-nous pu nous trouver dans une situation où le conseil de défense est devenu le lieu suprême de gestion de la crise sanitaire ? En vérité, l'objectif d'une telle manoeuvre a tout simplement été d'installer une gestion solitaire et autoritaire autour du Président de la République, qui a marginalisé le Gouvernement, les corps intermédiaires, le Parlement

Moi-même, je suis étonné qu'une institution dédiée à la défense nationale, à laquelle participent le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de chacune de nos armes, le chef d'état-major particulier du Président de la République, le secrétaire général de la défense nationale, le ministre de la défense, le Premier ministre ou encore le ministre des finances, et ayant vocation à prendre des décisions relevant de la stratégie de défense de la France puisse être réunie pour un sujet sur lequel les personnalités que j'ai mentionnées n'ont que peu de valeur ajoutée par rapport au ministre de la santé, au directeur général de la santé, au directeur général de l'offre de soins, au président de la Haute Autorité de santé, entre autres ... Et si l'on réunit ces personnes sans les militaires, ce n'est plus un conseil de défense. Mais, mes chers collègues, cette institution est placée sous l'autorité du seul Président de la République. Il en fait ce qu'il en veut. Je conteste formellement la pertinence de l'utilisation du conseil de défense pour gérer la crise sanitaire. Mais je ne vois pas comment le Parlement pourrait en quelque sorte faire intrusion

sont une formation spécifique du conseil de défense et de sécurité nationale, dont l'existence est prévue par l'article 15 de la Constitution. Ils permettent de réunir les membres du Gouvernement

un contournement du conseil des ministres ou du Parlement, qui ont, me semble-t-il, pleinement joué leur rôle depuis près de deux ans- notre débat de ce soir en témoigne -, notamment dans le cadre de l'examen des douze projets de loi relatifs à la gestion de la crise sanitaire. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

passé de façon totalement illégale puisque le refus de se soumettre à un test PCR a suffi pour envoyer en garde à vue un certain nombre d'étrangers, et pour les replacer ensuite en détention. Ces actes illégaux ont été contestés et la Cour de cassation a confirmé leur illégalité. Mais en août dernier, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, le Gouvernement a légalisé cette pratique en faisant voter un amendement visant à inclure dans le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Concrètement, un étranger qui refuse de se soumettre à un test PCR sera renvoyé en garde à vue et en détention. C'est indigne ! Cette mesure n'est en aucun cas une mesure sanitaire. Elle détourne les dispositifs de gestion de crise au service d'une politique migratoire inhumaine. S'opposer à un acte médical est une liberté fondamentale, que l'on refuse à ces personnes. Cette situation kafkaïenne a été pointée du doigt à de nombreuses reprises par des médecins, des universitaires ainsi que des associations engagées

Même avis.

est impératif de s'assurer que la règle du jeu permettra à tous les Français de voter. Je trouve que votre initiative, mon cher collègue, est excellente. Je regrette simplement qu'elle relève de la loi organique, ce qui nous empêche de l'adopter dès maintenant.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire quand il s'agit de sauver l'élection présidentielle, qui est la clé de voûte de nos institutions. Il y a une spécificité de cette élection : ainsi, la

Vous savez tous que ces élus et leurs représentants doivent être réellement et concrètement associés à toutes nos réflexions, et combien leur connaissance du terrain est nécessaire pour nous guider.

Il n'est nullement fait état dans la loi que le préfet « fait parvenir les mesures envisagées » pour faire face à l'épidémie, afin que les élus locaux et les parlementaires « puissent exprimer un avis sur ces dernières et faire des propositions ». Tel est le coeur du problème.

Le passe vaccinal est une mesure hautement coercitive et restrictive de libertés pour la population. Il convient que le Parlement, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, évalue la proportionnalité, l'utilité et les conséquences de cette mesure dans le cadre de la crise sanitaire, conformément au VI de l'article 1 de la loi du 31 mai 2021, qui prévoit que « l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, beaucoup de choses ont été dites sur cet article et, malgré tout, de nombreux malentendus persistent. Je souhaite donc clarifier nos objectifs et les raisons pour lesquelles nous souhaitons le rétablir. D'abord, contrairement à ce que j'ai entendu dire, il s'agit non pas de s'immiscer dans l'organisation des entreprises, mais de sanctionner les comportements de celles qui refusent délibérément de prendre les mesures de prévention nécessaires pour protéger la santé de leurs salariés face à la covid-19. Ensuite, j'entends parler de rupture de confiance, voire de suspicion généralisée. Dire que certaines entreprises ne jouent pas le jeu, cela n'est pas une rupture de confiance, c'est un constat C'est dire que la confiance que nous avons tous dans nos entreprises ne doit plus être entachée par les comportements dangereux de certaines. Comment peut-on affirmer que nous n'avons pas confiance dans les entreprises, alors que nous avons mobilisé des moyens sans précédent pour les protéger et les accompagner face à la crise ? C'est l'argent des Français ! Nous avons soutenu nos entreprises, coûte que coûte, depuis deux ans. D'ailleurs, bon nombre de chefs d'entreprise me disent qu'ils comprennent très bien, voire qu'ils appellent de leurs voeux, les sanctions prévues lorsque les obligations qui s'appliquent à tous ne sont pas respectées par certains. Par ailleurs, il faut redire qu'une procédure de sanction existe déjà. Nous cherchons à la rendre plus efficace, plus opérante, sans pour autant en changer l'esprit. Je rappelle que la procédure de sanction actuelle, tout comme celle qui vous est proposée, n'intervient qu'après une mise en demeure, ce qui laisse à l'entreprise un délai pour se conformer à ses obligations. Nous proposons une alternative à la procédure pénale en vigueur, laquelle aboutit dans un délai moyen de deux ans, ce qui n'est pas compatible avec l'urgence de la pandémie. Par ailleurs, nous faisons face à une question essentielle d'équité. Pour se conformer au protocole sanitaire, les entreprises doivent revoir leur organisation et acheter du matériel de protection. Tout cela représente, à la fois, des complications et des coûts pour l'entreprise. Comment pourrions-nous nous satisfaire, alors que la majorité des entreprises investissent autant de temps et d'argent, l'inverse, celles qui ne le font pas ne soient pas inquiétées ? Cela ne serait ni compréhensible ni juste. En supprimant tout simplement cet article, vous acceptez que certaines entreprises peu scrupuleuses jouent avec la santé des salariés et de leurs proches. Votre vote d'aujourd'hui renverra chacun à sa responsabilité ! Souhaitez-vous véritablement protéger l'ensemble des Français face à la crise, ou seulement l'ensemble des Français moins quelques-uns ? Pour conclure, je veux rappeler que l'enjeu, derrière ce débat, ce sont des vies. Il est de notre responsabilité de mettre en place les procédures nécessaires pour protéger tous les Français. Je vous invite à choisir la voie de la responsabilité en votant cet amendement.

de Roissy, des contrôles sont intervenus pendant huit mois d'affilée sans que l'entreprise se mette en conformité avec ses obligations. La situation ne s'est réglée

des dispositions permettant de sanctionner les entreprises qui ne font pas face à leurs obligations, et nous ne sommes pas d'accord avec cette nouvelle procédure, qui, à mon avis, perdurera bien après la crise sanitaire

Celles qui ne le jouent pas seront sans doute dissuadées de ne pas appliquer les protocoles.

Le maintien « quoi qu'il en coûte » de l'activité économique du pays au moment où le virus connaît une très forte circulation de doit pas nous empêcher de faire tout ce que nous pouvons pour protéger les Françaises et les Français. Les multiples hésitations et la frilosité du Gouvernement l'imposition d'un protocole sanitaire strict pour éviter les contaminations dans les entreprises ont conduit à un flou dans l'application des règles et des recommandations. Aujourd'hui encore, certains salariés se voient refuser la pratique du télétravail alors que cette dernière serait possible,

part d'une bonne intention, mais le dispositif prévu passait largement à côté de son objectif. La procédure d'instruction contradictoire précédant le prononcé d'une amende administrative est longue- elle aussi peut durer plusieurs mois.

Comment expliquer que les restaurateurs, les patrons de bar et de lieu culturel aient été transformés en douaniers sanitaires ces derniers mois, alors que les inspecteurs du travail, dont le métier est de protéger celles et ceux qui travaillent, se trouvent impuissants pour endiguer la propagation du virus dans les entreprises ?

pour toute ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'un service lorsqu'un ou plusieurs travailleurs ou travailleuses se trouvent dans une situation dangereuse avérée, en conséquence de l'insuffisance des mesures de prévention

identiques visent des situations beaucoup trop larges et trop difficiles à maîtriser pour les entreprises, même celles qui sont de bonne volonté, dans la mesure où l'exposition à un virus peut être généralisée. Le dispositif donne ainsi un pouvoir d'appréciation disproportionné à l'inspection du travail. La commission a donc considéré que les recommandations, les contrôles et les sanctions étaient déjà suffisants pour assurer la lutte contre la covid-19 au sein des entreprises, qui se sont largement mobilisées depuis le début de la crise.

Nous allons donc ouvrir la nuit afin de terminer l'examen de ce texte. Notre ordre du jour du jeudi 13 janvier prévoit, à partir de dix heures trente, l'examen de deux propositions de loi dans le cadre de l'espace réservé au groupe Union Centriste. En conséquence, si nous ne parvenions pas à finir l'examen de ce projet de loi cette nuit à une heure trente, nous devrions, en accord avec nos collègues de l'Union Centriste, décaler d'autant le début de cet espace réservé.

sociales ? Les entreprises sont déjà chargées d'évaluer les risques professionnels et de prendre les mesures qui permettent de prévenir ces risques, en concertation avec les salariés dans le cadre du dialogue social et sous le contrôle de l'inspection du travail.

de la crise, le Gouvernement cherche à concilier le maintien de l'activité des entreprises et la protection de la santé des salariés. C'est tout l'objet du protocole sanitaire en entreprise, qui vise précisément à définir les pratiques à mettre en place

Pour autant, contrairement à ce que j'ai pu entendre dire, le Gouvernement n'a pas à s'immiscer dans l'organisation des entreprises. C'est bien à l'employeur qu'il appartient, au titre de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité, de fixer, en associant les acteurs du dialogue social, les mesures d'organisation permettant de garantir la continuité de l'activité et la préservation de la sécurité des salariés. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

en faisant explicitement de cet état un cas de contre-indication médicale. En effet, si le passe vaccinal comme outil d'incitation à la vaccination ne peut être exigé au-dessous d'un certain âge- 16 ou 18 ans en fonction du dispositif retenu -, il est logique que les enfants à naître soient également exclus de cette vaccination, d'autant qu'il n'existe encore aucune étude de long terme concernant les effets potentiellement indésirables du vaccin

incombe aux autorités de santé indépendantes de formuler les recommandations en matière de vaccination. Ensuite, sur le fond, cette disposition laisse entendre que le vaccin pourrait être dangereux pour les femmes enceintes, qui constitueraient un public à risque. Or c'est exactement l'inverse, puisque les femmes enceintes sont considérées comme prioritaires pour la vaccination. En particulier, le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale

un risque majeur d'être césarisée en urgence. C'est ce qui s'est produit dans plusieurs hôpitaux, en particulier à Bichat, pour des mamans vraiment très mal en point. Et je ne développe même pas le cas des futures mamans en réanimation, où le risque est de perdre et la maman et le bébé. Il faut vacciner les femmes enceintes

de cet amendement, de ne pas inciter à la vaccination de femmes qui sont à haut risque de complications, pour elles-mêmes et pour leur bébé.

est à Mme Laurence Cohen. Le droit du travail est guidé par un certain nombre de principes fondamentaux, qui font office de garanties pour les salariés, lorsque ces derniers sont confrontés au risque de perte de leur emploi ou de leur rémunération.

rupture dudit contrat, d'un revenu de remplacement ou d'allocations sociales. Cette politique constitue l'un des piliers de l'État providence, garantissant à chaque individu un minimum de ressources pour subsister et conserver une certaine dignité. Tous ces droits

Si sanction il doit y avoir, celle-ci ne saurait être aussi disproportionnée, car cela conduit au placement brutal d'un certain nombre de salariés dans une situation de précarité sans précédent. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons revenir sur cette disposition,

Cet amendement vise donc à permettre le retour des non-vaccinés, en revenant à la situation antérieure au 15 octobre 2021, ce qui permettait aux non-vaccinés de travailler sur présentation d'un test de dépistage. s'appliquerait aux personnes soumises à l'obligation de vaccination en vertu de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, qui inclut les soignants, mais également les pompiers et les transports sanitaires. L'amendement

de Mme Muller-Bronn tend à permettre aux professionnels soumis à l'obligation vaccinale de continuer à exercer leur activité

L'amendement n° 145 de Mme Assassi est similaire à celui de Mme Jasmin, que j'ai

quand on voit la difficulté qu'il y a à convaincre la population de se faire vacciner et le manque de personnel hospitalier, on se dit que l'on marche sur la tête.

En Bretagne, par exemple, les entreprises de transport cherchent 540 chauffeurs. Il est donc indispensable, à mon sens, que l'on prenne des dispositions

sociales, il s'agit d'une mesure de justice en faveur des retraités qui participent à l'effort collectif pour soutenir l'ensemble des soignants épuisés depuis

éviter toute rupture de trésorerie, à sécuriser les financements des établissements et à leur donner une visibilité budgétaire pour assurer pleinement la prise en charge des patients,

Mme la ministre déléguée. Cet amendement vise à rétablir l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires au bon fonctionnement des copropriétés,

plus que l'accumulation des reports de rendez-vous s'avère préjudiciable pour l'organisation des entreprises et pour les travailleuses et les travailleurs et que les SST peuvent aider à convaincre, lors desdits rendez-vous, les salariés non encore vaccinés. La médecine du travail, investie d'une mission d'ordre public social, doit préserver ses prérogatives. Il est indispensable de la laisser effectuer ses missions quotidiennes, qui touchent des enjeux divers, en lien avec la pénibilité du travail, la prévention du harcèlement moral et sexuel au travail, le maintien dans l'emploi des travailleurs ou encore l'ergonomie des postes de travail.

la ministre déléguée. Cet amendement vise à permettre de prolonger les dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales au bénéfice des employeurs et travailleurs indépendants les plus touchés

Le déploiement d'autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 par prélèvement nasal ne nécessite pas la présence de professionnels de santé, ce qui permet la réalisation de tests plus fréquents au sein de la population. Il s'agit d'un outil essentiel dans la lutte contre le virus. Il est donc indispensable d'augmenter les disponibilités de ces tests et d'en permettre l'accès au plus grand nombre. Les auteurs de cet amendement proposent de pérenniser les mesures mises en place par l'arrêté du 27 décembre 2021

Les pharmaciens sont des professionnels de santé ; ce ne sont pas des épiciers qui se contentent de délivrer des médicaments ou des dispositifs médicaux. Ils apportent

J'espère ne pas avoir à subir la furie, voire la fureur, du tribunal révolutionnaire de la République vaccinale ... Permettez-moi de dénoncer ce qu'il s'est passé voilà quelques

la manière dont notre collègue a été traitée pour avoir commis le crime de présenter un amendement visant à exempter les femmes enceintes de l'obligation vaccinale. Personne ici n'est antivax ; en revanche, il est des sénateurs qui sont contre l'obligation vaccinale. Pour avoir présenté cet amendement, notre collègue a été montrée du doigt.

Le ministre Véran nous demandait hier de croire à la science : je suis, pour une fois, totalement d'accord avec lui. Le port du masque dans la rue est inutile : il ne fait qu'accentuer la séparation des Français et alimenter la psychose. Il est temps de s'en débarrasser.

d'empêcher une telle mesure. Par ailleurs, cette obligation est très encadrée. Le Conseil d'État a précisé, dans une ordonnance du 11 janvier dernier, que les préfets ne peuvent imposer le port du masque en extérieur qu'à certaines

Aussi, notre groupe propose d'imposer une protection plus grande pour la population dans les transports publics collectifs, où les gestes barrières de distanciation et d'aération sont parfois totalement impossibles. Cependant, les FFP2, plus protecteurs, sont plus chers que les masques chirurgicaux, dont le coût pèse déjà beaucoup sur les budgets des ménages.

sans filtre dans les établissements recevant du public et dans les transports en commun, qui sont, chacun ici le sait, des lieux à haute contamination.

installations aux collectivités, alors que cette mesure de bon sens devrait figurer au coeur de la stratégie de lutte contre l'épidémie du Gouvernement. L'installation de détecteurs de CO2 est pourtant la mesure la plus simple et la moins coûteuse pour contrôler la qualité de l'air. Ces capteurs contribuent à lutter contre la propagation du virus, la concentration de CO2 permettant de s'assurer que les salles sont suffisamment aérées. Ils peuvent également devenir un outil pédagogique, qui permet de sensibiliser les enseignants, les enfants, mais aussi les parents au réflexe de l'aération des pièces. En France, certaines régions et villes commencent à se doter, sur leur propre budget, de cet équipement,

Mme la rapporteure

maires, les présidents de département et les présidents de région, expliquez-leur le dispositif d'accompagnement du Gouvernement pour équiper les écoles, de la maternelle à l'université, avec des capteurs de CO2 et des purificateurs. La

En effet, le 1décembre dernier, lors de l'audition devant la commission des affaires sociales du Sénat, différents agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont pu s'exprimer sur les effets indésirables faisant suite à l'injection des vaccins ARN anti-covid.

un rapport actualisé de pharmacovigilance sur les vaccins et les traitements. La commission des affaires sociales a auditionné en décembre dernier

toutes les tranches d'âge, le taux de vaccination dans les communes et les quartiers les plus défavorisés reste significativement inférieur à celui qu'on observe dans les communes les plus favorisées.

Ses conclusions devront permettre d'accélérer la vaccination, ce qui est le but du Gouvernement et de la plupart d'entre nous, auprès des populations les plus fragiles et les plus isolées et de présenter un bilan des actions prises, afin qu'elles ne viennent pas s'ajouter à des fractures préexistantes. l'avis de la commission ses compétences de contrôle de l'action du Gouvernement, que nous entendons régulièrement, tout comme les autorités sanitaires, l'assurance maladie ou le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

commission des affaires sociales de travailler et d'auditionner ces organismes.

sauf pour raison médicale, les tests de dépistage de la covid-19 sont tous devenus payants pour les adultes non vaccinés. Les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance doivent débourser la somme minimale de 44 euros pour un test PCR, 22 euros pour un test antigénique en laboratoire, 25 à 30 euros en pharmacie, 5,20 euros pour un autotest et 12,90 euros s'il est supervisé par un professionnel de santé. Ce budget peut être important pour les personnes en situation de précarité. Plusieurs conséquences prévisibles ont été constatées sur cette catégorie de population, en particulier une baisse du taux de dépistage pour les adultes non vaccinés et une baisse de dépistage pour les adultes asymptomatiques.

il paraît nécessaire de revenir sur cette mesure, afin que l'ensemble des Français puissent avoir recours à un dépistage non conditionné à leurs moyens financiers. l'avis de la commission je voudrais revenir sur un point de votre amendement. Vous parlez en effet de « gratuité ». Or la gratuité n'existe pas, vous savez bien que c'est pris en charge par l'assurance maladie. Ce n'est pas tout à fait la même chose de dire que c'est « gratuit

soit prise en charge par les départements, dans des conditions qui leur donneraient vraiment les moyens de la mettre en place. Madame la ministre, selon moi, la crise sanitaire montre l'enjeu

Nous aurons à débattre prochainement d'un texte sur le harcèlement scolaire. Là encore, la médecine scolaire est forcément

au commerce, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Une telle dérogation faciliterait le partage de la propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaire pour accroître et accélérer la disponibilité, l'accessibilité et le caractère abordable des vaccins, tests et traitements contre la covid-19 dans le monde. le monde. En 2001, sous la pression de l'opinion publique mondiale, les laboratoires pharmaceutiques avaient finalement dû se résoudre à laisser l'Afrique du Sud, ravagée par l'épidémie de Sida, faire produire en Inde des génériques d'antiviraux. Ce fut un véritable tournant dans l'histoire des À l'époque, il s'agissait de permettre la fabrication de génériques de synthèse. Aujourd'hui, accéder au brevet de ces vaccins de nouvelle génération reste insuffisant. La déclaration commune lancée sur l'initiative de Médecins sans frontières, qui sera rendue publique ces prochains jours, insiste également sur l'accès « au savoir-faire, aux données et aux ressources » liées à la recherche et développement. L'enjeu est tel qu'il nécessite un engagement majeur des États auprès des institutions internationales pour que les laboratoires acceptent de transférer les technologies développées. Signataires de cette déclaration commune, les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaitent que la France soutienne activement cette position au niveau international,

des affaires sociales ? L'objet de cet amendement a été abordé à plusieurs reprises, en particulier lors de l'examen de l'article 1. du partage des droits pour la recherche, l'accès et la production du vaccin va bien au-delà des cadres national et européen. Les différentes firmes et les différents laboratoires

Mme la ministre déléguée. Cet amendement vise à rétablir les possibilités offertes par l'ordonnance du 25 mars 2020 aux assemblées et aux organes dirigeants des personnes morales et autres entités de droit privé en matière de réunion et de délibération à distance, ces dispositions étant arrivées à échéance en septembre 2021. Dans le contexte actuel de reprise de l'épidémie, il s'agit, d'une part, de permettre au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures nécessaires au bon fonctionnement des réunions et des délibérations de ces entités et, d'autre part, d'autoriser immédiatement les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, par exemple les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés, à se réunir et à prendre des décisions à distance.

Nous nous sommes dit néanmoins que, plutôt que d'émettre un avis défavorable pour une raison juridique, nous pouvions nous en remettre à la sagesse de notre assemblée.

Nous n'avons pas le pouvoir de le sortir de cet embarras ; croyez bien, madame la ministre, que je le regrette profondément. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Ce dispositif a permis aux organisateurs de manifestations culturelles et sportives contraints d'annuler leurs contrats de vente de billets et d'abonnements du fait de la crise de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées.

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité que les prestations de serment réalisées au cours d'une audience juridictionnelle soient faites par écrit. Cette possibilité évite les rassemblements de nombreuses personnes venant ensemble prêter serment, nouveaux auditeurs reçus à l'École nationale de la magistrature, élèves avocats et nouveaux avocats, etc. Elle est donc un outil nécessaire à la lutte contre la propagation de la pandémie.

en breton.

contexte n'est plus à établir. Les dispositions supprimées par la commission des lois ont vocation à permettre un nouvel usage, essentiel, des données qui y figurent, en ajoutant aux finalités des systèmes d'information destinés à la lutte contre la covid-19 le contrôle du respect de l'obligation de dépistage par les personnes mises en quarantaine ou en isolement

des SI covid-19 sera donc très circonscrite dans son objet. Les dispositions proposées ont été jugées conformes aux règles de protection des données par le Conseil d'État, dans l'avis qu'il a rendu sur ce projet de loi. Elles seront précisées par décret

C'est là une position constante du rapporteur et de la commission. Toutefois, il me semble que dans un cas précis,

? Ce sujet est complexe et assez spécifique. Il y a des mises à l'isolement de personnes qui viennent de l'étranger et sont malades et il y a des mises en quarantaine de personnes qui viennent de l'étranger et sont simplement cas contact. Isolement, quarantaine, ce n'est pas tout à fait le même régime ... Il n'est pas prévu, dans les textes, de test de dépistage pour sortir de l'isolement ou de la quarantaine. L'obligation qui serait faite

cet article vise à combler une double censure du Conseil constitutionnel, triple censure, même, puisque le Gouvernement, malgré les avertissements du Sénat, avait inscrit au projet de loi de financement de la nous nous retrouvons à devoir adopter en urgence une disposition qui requiert une particulière vigilance dans un véhicule législatif- disons-le -peu approprié. Une question, ensuite, liée à cette urgence, justement. Depuis le 1 janvier 2022, les dispositions relatives au renouvellement des mesures d'isolement et de contention sont abrogées.

Mes questions sont donc simples : quelle est la situation concrète dans les services de soins sans consentement depuis treize jours ? Comment de telles mesures d'isolement ou de contention sont-elles prises et renouvelées ? Comment les médecins et hôpitaux sont-ils en capacité de veiller à la sécurité des patients, mais aussi de leur environnement et des soignants ? Le juge est-il en mesure d'être saisi et de faire respecter les droits fondamentaux des patients ? La parole

la rapporteure pour avis, à la double décision du Conseil constitutionnel, qui ordonnait une révision de la loi avant le 31 décembre 2021. La date passée, nous nous trouvons face à un vide juridique. En conséquence, les mesures d'isolement et de contention ordonnées ordonnées depuis le 1 janvier n'ont plus de cadre légal. Mais on ne peut contester que cet article ne présente aucun lien, direct ou indirect, avec le texte de loi que nous examinons.

nationale prouve, s'il était nécessaire, que le débat fondamental sur ces dispositions n'a pas eu lieu et risque dès lors d'être forclos pour très longtemps. Ce faisant, la psychiatrie reste le point aveugle de nos débats sur la santé, comme la psychiatrie est le parent pauvre de l'Ondam. Pourtant, l'audition de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a montré l'urgence d'un débat sur l'usage, voire le mésusage, des pratiques de contention et d'isolement et l'exigence d'explorer de possibles alternatives.

en psychiatrie depuis le 1 janvier. Compte tenu des effets à compter de cette date de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021 et de la censure de la réforme que nous avions proposée dans le cadre du PLFSS pour 2022 pour tirer les conséquences de cette décision,

ne peut légalement être maintenue au-delà des durées respectives de quarante-huit heures et de vingt-quatre heures. En conséquence, aucune disposition législative ne permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de ces mesures au-delà de ces durées. Cette limitation dans le temps des mesures d'isolement et de contention n'a pas pour effet de priver le juge des libertés et de la détention de sa compétence à contrôler lesdites mesures, les dispositions afférentes demeurant en vigueur. En complément, je dois dire que, dans le contexte déjà difficile qui est celui de la psychiatrie- pénurie de psychiatres et d'infirmiers, nombre croissant de malades -, cette censure complexifie le quotidien des équipes soignantes alors même qu'un texte d'équilibre avait été trouvé entre les représentants des patients et les représentants Les dispositions prévues par l'article 3 permettront de remédier à cette situation transitoire et j'espère, à cet égard, que ce projet de loi pourra être promulgué dans les meilleurs délais.

revanche, sur le fond, vous avez tout à fait raison : cet article n'a strictement rien à voir avec la crise sanitaire. Et le véhicule législatif retenu n'est pas forcément, loin de là, le plus pertinent. Pour autant, son adoption est sans doute tout aussi urgente que celle de l'article 1, dont l'effet est attendu dès l'instauration du passe vaccinal. En effet, l'article 3 vise à combler le vide juridique qui prévaut depuis le 1 janvier 2022,

aux fins de mainlevée de la mesure ». Nous l'avions souhaité nous aussi ; nous nous en réjouissons. Nous constatons cependant que cette référence ne mentionne pas explicitement la personne de confiance la personne de confiance instituée par la loi de 2002, dont les missions ont été précisées par la loi de 2016. Or celle-ci s'avère particulièrement utile en pareille situation. Un article du code de la santé publique précise que « lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé [ ...], il est proposé au patient de désigner une personne de confiance », dont le rôle est d'accompagner le patient dans ses démarches de l'aider à prendre des décisions. Cette personne doit être associée à la recherche du consentement du patient. Cette personne, si elle a été désignée, doit en conséquence être informée lorsqu'est prise une mesure d'isolement et de contention. Dès lors, en cohérence avec le code de la santé publique et dans un souci de respect de l'intérêt et des droits des patients, il nous semble pertinent d'ajouter nommément à la liste des personnes informées visée à l'article 3 la

nos amendements ont été suggérés par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui a trop souvent constaté des conditions matérielles d'isolement méconnaissant le respect de : lieux indignes, absence d'accès à l'eau ou à des sanitaires, absence de bouton d'appel, matelas directement posés sur le sol, intérieurs de chambres visibles par les autres patients, etc.- il arrive même que Le juge ne doit donc pas seulement vérifier la réalité de l'existence des conditions qui justifient la mesure- danger pour le patient ou pour autrui -, mais également que la mesure ne porte pas atteinte à la dignité et à l'intimité de la personne.

Dans son rapport sur cette question, en 2017, la Haute Autorité de santé soulignait que les mesures d'isolement et de contention doivent toujours « respecter les droits des patients à la dignité et au respect de leur intégrité corporelle »,

si l'on en juge par les nombreux signalements pour traitements dégradants- ma collègue vient d'évoquer ce point -relevés par les autorités depuis des années. En 2016 et en 2020, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté rendait ainsi deux rapports accablants sur les conditions de prise en charge des patients en psychiatrie.

sociales ? Ces amendements nous semblent satisfait. En effet l'article L. 1110 -2 du code de la santé publique prévoit déjà que la personne malade, quel que soit son état,

Le placement en soins sans consentement de tels patients ne correspond pas aux conditions prévues par la loi de 2011. Or le changement de statut d'admission entraîne des conséquences juridiques particulièrement graves, qui ne sont pas justifiées par l'état clinique

justifié. Rappelons que le délai de six heures tient compte également des temps de changement d'équipe, qui peuvent influer sur l'évolution du patient. Enfin, il faut ajouter que si, en situation de crise, il est nécessaire de pratiquer une contention concomitante à l'isolement, le même délai de six heures reste cohérent avec le délai de six heures de la contention prévu dans le texte en discussion. Quel est l'avis de la commission

Mme Raymonde Poncet Monge. Je l'ai dit et je le répète, car c'est important : le code de la santé publique affirme le caractère de « dernier recours » de l'isolement et de la contention. Toutefois- Laurence Cohen l'a signalé -, le manque de personnel, conjugué aux insuffisances chroniques de financement des soins en psychiatrie et à d'autres conditions organisationnelles dégradées, conduit trop souvent le personnel de certains établissements à recourir aux mesures d'isolement et de contention, au risque de porter atteinte aux droits fondamentaux des patients. Dans son commentaire sur sa visite récente au centre hospitalier du Forez, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté

À ce constat alarmant s'ajoutent de vives interrogations quant à l'intérêt thérapeutique des mesures d'isolement ou de contention. Selon le Conseil de l'Europe, effet, « il convient de reconnaître que le recours à des mesures de contention semble être influencé de manière non négligeable par des facteurs non cliniques ». De nombreuses voix s'élèvent désormais pour proposer des alternatives à des mesures qui comportent effectivement, quasi intrinsèquement, des risques de dérives. Certes, il faut combler le vide- et le présent amendement vise à en souligner l'urgence -, mais nous ne pouvons accepter l'absence d'un débat sur les mesures d'isolement et de contention.

punitive de contraintes, nous refusons cette latitude trop grande accordée au pouvoir exécutif dans la détermination et dans l'application, dans le temps, de mesures restrictives et liberticides. Nous ne voterons donc pas ce texte. Je lui transmettrai

en affirmant que les libertés étaient sacrées, mais qu'elles n'étaient pas absolues, se faisant ainsi et se faisant encore le rapporteur de l'Élysée. Quand les moyens choisis sont adaptés, nécessaires et proportionnés en vue du bien commun, chacun peut accepter de restreindre sa liberté. Ce fut le cas lors du premier confinement. Mais dix-huit mois se sont écoulés, mois d'analyses scientifiques, qui démontrent les mêmes incidences contagieuses chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Et pourtant vous vous obstinez. Ensuite, M. le rapporteur a ajouté que la liberté consistait à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Si je traduis, les non-vaccinés sont nuisibles.

ce sont ceux qui ont plongé l'hôpital dans la détresse, par des suppressions de postes, par les 15 000 suspensions de personnels soignants non vaccinés et par des fermetures de lits par dizaines de milliers. Votre rigueur budgétaire a tué la rigueur sanitaire. C'est cette folie que, tous, vous voulez masquer, quitte à martyriser les libertés des Français. Comme le chef de l'État candidat, vous voudriez que l'arbre de la covid puisse cacher votre funeste bilan. Adopter ce passe vaccinal, c'est accepter la logique du passe dans tous les domaines de la vie : passe sanitaire, passe vaccinal, passe électoral, passe écologique ! Nos libertés trépassent l'examen de ce texte, et malgré toutes vos gesticulations, vous fermez les yeux devant la disparition durable de nos droits et de nos libertés fondamentales, en votant sous le coup de la peur et non sous la conduite de la raison, un passe vaccinal qui n'aura aucun effet sur l'épidémie de covid-19. Alors j'en appelle directement aux Français. Que l'évidence et la providence les guident pour s'administrer, le moment venu, le vaccin électoral qui les soulagera de ceux qui auront insulté et divisé le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Quant à moi, je voterai de toutes mes forces contre ce texte les intentions de ses auteurs.

Nous avons entendu la promesse de ne jamais rendre la vaccination obligatoire, celle de ne jamais généraliser le passe sanitaire aux actes de la vie courante, puis celle de ne jamais transformer ce passe en